mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je suis heureux de saluer la présence dans nos tribunes des auditrices et auditeurs de la septième promotion de l’Institut du Sénat, accueillie hier par la vice présidente Sylvie Robert. Sur l’initiative de notre

en vue de mieux faire connaître les modalités de fonctionnement et les enjeux de notre démocratie parlementaire à des personnalités d’horizons géographiques et professionnels très divers. neuf auditeurs de la septième promotion, issus de dix départements et de trois organismes nationaux différents, représentent en effet des sphères d’activités professionnelles, publiques, éducatives, juridiques, scientifiques, médicales, économiques, ou

En votre nom à tous, je leur souhaite une excellente session au Sénat. Je suis certain que, à l’issue de leur mission de quatre mois, ils pourront être les témoins privilégiés de la place essentielle de notre institution au sein de la V République et de la qualité du travail parlementaire.

rurale (ZRR) et la mise en place du dispositif France Ruralités Revitalisation (FRR) n’en finissent pas de susciter des interrogations et des craintes sur notre territoire. Certes, un accord a été validé en loi de finances, ici, au Sénat, après de longs débats budgétaires. Toutefois, les données dont nous disposions ne nous permettaient pas d’objectiver l’impact d’une telle réforme sur nos territoires.

tout particulièrement notre attention. Je le redis avec force et conviction : je suis à votre entière disposition pour que nous trouvions la solution la plus adaptée à chacune de nos communes. La parole

Monsieur le ministre, à quelques jours du vote au Sénat du projet de loi autorisant la ratification de deux accords entre l’Union européenne et le Canada, ma question s’adresse à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et concerne la défense de la souveraineté maritime de la France en Amérique du Nord. La ratification de ces accords, sans réserve formelle de la part de la France, risquerait de constituer un abandon de toute défense de nos intérêts maritimes dans cette zone, au profit du seul intérêt économique. Dans son article 1.3, l’accord

Concernant le plateau continental, les demandes d’extension de la France et du Canada déposées aux Nations unies concernent une zone commune qui,, nécessitera un accord entre ces deux pays, dans un cadre de respect mutuel. Cette question est d’autant plus urgente que l’archipel de Saint Pierre et Miquelon attend la concrétisation des engagements pris par le Gouvernement lors de l’examen du Ceta – l’accord économique et

Ces accords ne peuvent ni constituer une reconnaissance de la ZEE canadienne ni un abandon par la France de ses demandes devant les Nations unies. Face à ces enjeux urgents, ma question est simple. La France défendra t elle ses deux réserves pour préserver ses intérêts en Amérique du Nord ? ? Le Gouvernement créera t il enfin le fonds promis depuis 2019 en faveur de Saint Pierre et Miquelon pour asseoir le rayonnement de la France dans cette partie du monde ? La parole

La parole est à Mme Marie Pierre Monier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

On l’accuse d’islamophobie alors qu’il se bat pour ses élèves, dénonce la ghettoïsation des établissements scolaires. […] Cela doit être douloureux pour lui. » Le déroulement des faits, glaçants, nous en rappelle d’autres, qui ont conduit au pire.

ils font état d’un climat de tensions sans précédent et d’une peur au ventre qui les taraude. Les chiffres publiés par le ministère de l’éducation nationale témoignent d’une hausse du nombre d’incidents graves.

Notre pays compte plus de 5,2 millions de passoires thermiques. Il y fait trop chaud l’été, ou bien trop froid l’hiver, et le gaspillage énergétique induit est coûteux tant pour les résidents que pour la planète et même insupportable pour les plus précaires. La rénovation de ces logements est une urgence d’un point de vue écologique, social et économique. Tous les acteurs sont concernés : les bailleurs, qu’ils soient privés ou sociaux, et les professionnels du bâtiment, qui voient dans les chantiers de travaux de rénovation une façon de compenser le manque de constructions neuves, problème que vous ne traitez pas.

Vous dites avoir à cœur de ne pas laisser les finances publiques dériver. Tous les scientifiques le disent pourtant déjà : le coût de votre inaction sera bien supérieur lorsqu’il faudra faire face aux dégâts du dérèglement climatique, contre lequel vous n’agissez pas. Parmi les plus de 12 millions de personnes vivant dans un logement mal isolé, qui laisserez vous dans la précarité ? Parmi les bâtiments qui émettent 64 millions de tonnes de CO2, lesquels laisserez vous encore dégrader le respect de nos objectifs écologiques ?

aux économies budgétaires qui sont nécessaires dans un contexte difficile sur le plan des finances publiques. Nous avons donc accepté de renoncer à 1 milliard d’euros d’augmentation sur celle de 1,6 milliard qui était

Engendré par les alternances de pluies intenses et de sécheresses, il menace plus de dix millions d’habitations métropolitaines. Le Sénat a été le premier à se mobiliser contre les RGA. Dès 2019, nous avons mené une mission d’information sur le sujet, qui s’est traduite deux ans plus tard par l’adoption de la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, dont j’ai eu l’honneur d’être corapporteur. Cette réforme est elle aboutie ?

Les conséquences sont catastrophiques pour les habitants des communes déboutées, qui ne peuvent plus solliciter leur assurance habitation pour prendre en charge les dégâts – on parle de foyers ruinés et de vies brisées. En 2022, la Cour des comptes a pointé du doigt cette insuffisante prise en considération des réalités locales. Le député Vincent Ledoux a récemment présenté des propositions pour corriger ce dispositif. Ma question est simple

français en 2023 et a conclu que l’avancement du design du projet ne permettait pas à EDF de passer à la phase de design avancée sur certains bâtiments. Dans ce contexte,

pour assurer à terme des économies d’échelle. Dès réception du nouveau chiffrage par EDF, nous reviendrons bien évidemment devant la représentation nationale pour vous en rendre compte. Selon vous, le nucléaire est une « pompe à fric » ; pour nous, c’est une question de souveraineté nationale et d’investissement pour la Nation – ne négligeons pas l’intérêt national

Monsieur le Premier ministre, quelle différence votre gouvernement fait il entre une croix et une flèche ?

Non, madame la ministre, je le regrette, il ne s’agit pas de la même chose. Vous pouvez peindre la tour Eiffel dans la couleur que vous souhaitez, mais vous ne pouvez pas enlever la croix du dôme des Invalides, qui trône depuis Louis XIV.

Faites la Nation, toute la Nation ; la République, toute la République ; la France, toute la France ; n’effacez pas nos symboles

et indépendants. Ma question s’adresse à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Madame la ministre, je souhaite vous faire part d’une grande inquiétude liée au mouvement de protestation des producteurs de canne à sucre de mon territoire, la Guadeloupe. J’associe à cette question mon collègue Dominique Théophile. Les producteurs de canne sont à bout, pénalisés par la baisse des tonnages, l’augmentation du prix des intrants et la diminution de la richesse en sucre ; ils ne parviennent plus à couvrir leurs charges ni à tirer un revenu décent de leur exploitation.

Faisons d’abord supporter cet effort par le seul usinier encore présent en Guadeloupe et qui se trouve ainsi en position de force par rapport aux producteurs. Comment comprendre que le modèle de fixation des prix de la canne datant de plus de cinquante ans ne tienne compte que de la richesse en saccharine ? Les produits dérivés de la canne sont pourtant vendus très cher sur le marché international, générant pour l’usinier des revenus substantiels 5 millions d’euros de bénéfices et 16 millions d’euros de report à nouveau. Comment accepter que ces revenus ne soient pas redistribués aux producteurs ? Enfin, madame la ministre, comment comprendre que cet usinier soit habilité à distribuer les subventions européennes aux producteurs ? Il s’agit d’un moyen de pression La filière de la canne à sucre est en profonde souffrance ; il est temps d’arrêter de casser du sucre sur le dos des producteurs. Ceux ci iront jusqu’au bout de leur combat et ils peuvent compter sur moi pour porter ici leur voix.

Comme vous le savez, une convention sous l’égide de l’État régit les relations entre l’industriel et la filière canne en Guadeloupe. Cette convention, renouvelée il y a un an pour la période 2023

et par l’État de l’équivalent du net, revenant à 9 euros par tonne produite. Compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontés les planteurs, nous travaillons à de nouvelles avancées et des discussions sont en cours sous l’égide du préfet pour trouver un nouveau point d’équilibre entre les planteurs et l’industriel. Deux pistes

dès la campagne 2024 permettant la valorisation de tous les coproduits de la canne et conduisant à un meilleur partage des bénéfices. Pour autant, madame la sénatrice, pour que ces propositions aient du sens, il est impératif que la campagne de 2024 démarre. La collecte en temps et en heure de la canne est la garantie d’une richesse en sucre optimale et donc d’une meilleure rémunération des planteurs. Par ailleurs, au delà des prix, les discussions doivent porter sur le redressement de la production et des rendements à l’hectare. Il

Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, permettez moi de vous narrer un mauvais vaudeville en quatre actes. Acte I, 25 novembre, Sénat. La Haute Assemblée adopte en séance publique quatre amendements identiques au projet de loi de finances pour 2024, ainsi le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui des locations nues. Acte II, 16 décembre, Assemblée nationale. Le Gouvernement engage sa responsabilité. La loi de finances est adoptée. Surprise : elle maintient dans son article 45 les dispositions introduites par le Sénat. « Par erreur », affirme le Gouvernement. « Trop tard ! », lui répond la loi. Acte III, 29 décembre, palais de l’Élysée. Le Président de la République promulgue la loi : le régime fiscal des meublés de tourisme est aligné sur celui des locations nues. Telle est la loi. Acte IV, 14 février,. En contradiction avec la loi, le Gouvernement autorise les contribuables à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions du code général des impôts dans leur version antérieure

puisque les députés du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale n’ont pas voté cette proposition de loi et ont refusé un rééquilibrage des règles du DPE, de la fiscalité locative et des outils que nous souhaitons accorder aux élus locaux.

Monsieur le ministre, votre non réponse à ma question m’offre un formidable épilogue. 6 mars, Sénat : des explications confuses, mais si symptomatiques d’une méthode artisanale, doublée d’une petite dose de cynisme et de beaucoup d’arrogance. Telle est la chronique, devenue banale, d’un exécutif vacillant, piétinant sans vergogne le Parlement. Pendant ce temps, cinq ministres du logement se sont succédé en sept ans, mais aucune grande loi sur le sujet, pourtant maintes fois promise, n’a été adoptée. Voilà une parfaite illustration de l’absence de boussole de ce gouvernement, alors que sévit dans le pays une terrible crise du logement. Sur ce sujet crucial, moins de basses manœuvres, plus d’action : il y a urgence

Madame la secrétaire d’État, vous savez bien sûr qui est l’auteur de cette déclaration faite en 2022 : « Personne n’a envie que ses données de santé soient répandues aux personne n’a envie que les données de fabrication d’un Airbus, d’un TGV, d’un satellite ou d’Ariane soient diffusées à travers la planète. » Chacun, et vous la première, aura reconnu la plume du ministre de l’économie, dans ses œuvres complètes. Pour ces mots ne sont ils que des mots ? Il y a trois semaines était publié un article du selon lequel EDF aurait confié la planification de la maintenance de ses centrales nucléaires à Amazon, un Gafam, dans le cadre d’un contrat de 860 millions d’euros. Cette affaire est sérieuse et ne souffre ni caricature ni légèreté. Madame la secrétaire d’État, si cette information est fausse, pourquoi avoir attendu qu’une question soit posée à l’Assemblée nationale pour que votre collègue, M. Lescure – ici absent –, la démente du bout des lèvres ? Si elle n’est que partiellement fausse, veuillez nous indiquer avec précision dans quelle proportion : périmètre du marché, montant, objet précis. Si elle n’est que partiellement vraie, cela reste très grave. La représentation nationale veut maintenant des réponses précises, car l’unique actionnaire d’EDF, c’est nous, c’est l’État, et l’unique responsable, c’est vous

ou public. Comme l’a assuré EDF au Gouvernement, plusieurs expérimentations ont été lancées dans le cadre d’un programme de rénovation, dont une sur les pièces de rechange utiles au fonctionnement normal des centrales nucléaires. C’est à cette occasion que l’entreprise a fait appel au public d’Amazon Web Services

le d’AWS, les données confidentielles des centrales nucléaires d’EDF sont, par ailleurs, hébergées dans des infrastructures privées que l’entreprise gère en propre. Votre question, toutefois, monsieur le sénateur, relève d’une préoccupation majeure, que nous partageons : les entreprises stratégiques ont encore très insuffisamment recours aux offres de de confiance. Je souhaite donc réaffirmer que la doctrine de l’État est bien de veiller à ce que les données sensibles des administrations et des entreprises soient hébergées dans des infrastructures bénéficiant de la qualification SecNumCloud. La France est d’ailleurs engagée dans les négociations du futur schéma européen de certification des services de, l’EUCS (). Enfin, dans le cadre de France 2030, le Gouvernement mobilise 700 millions d’euros pour accompagner les acteurs dans cette labellisation SecNumCloud. Vous pourrez compter sur notre mobilisation, monsieur le sénateur, non seulement dans le suivi de ce dossier très précis, mais aussi pour faire appel aux leviers de financement nécessaires à l’émergence d’un marché français et européen compétitif d’offres de de confiance. Ce n’est

Trois semaines plus tard, vous entretenez toujours le flou, même si vous nous avez un peu renseignés sur le périmètre et la sensibilité des données. Nous ne savons toujours pas s’il s’agit d’une expérimentation et nous ne connaissons pas le montant

de la souveraineté alimentaire, en mai 2022, l’Union européenne décidait, par solidarité avec l’Ukraine, de lever les droits de douane et les quotas pour les produits agricoles ukrainiens. Deux ans plus tard, la concurrence de ces importations est devenue insoutenable pour nos agriculteurs. Sur le seul mois de janvier 2024, un million de tonnes de blé tendre ukrainien ont été importées en Europe, soit la totalité du volume par an avant la guerre ; le cours du maïs a également chuté de 30 %. Face à cet afflux devenu hors de contrôle, il est urgent que la Commission européenne réagisse. Dans sa proposition de règlement sur les échanges avec l’Ukraine, elle introduit, certes, un frein d’urgence pour les œufs, le sucre et la volaille, permettant de rétablir les droits de douane si les importations de ces produits dépassent un certain contingent annuel, mais elle oublie d’y inclure les céréales. Le Premier ministre a affirmé le 1 février vouloir engager une négociation à Bruxelles pour limiter les importations de céréales. Or les représentants de la France à Bruxelles ont voté le 21 février dernier en faveur de cette proposition, sans demander l’inclusion d’une clause de sauvegarde pour les céréales. La position de la France est incompréhensible. Êtes vous favorable ou non au déclenchement de la clause de sauvegarde pour préserver nos producteurs de blé et de maïs ? Quelles consignes allez vous donner à vos députés européens pour le vote du 7 mars prochain ?

est un soutien résolu de l’Ukraine, car défendre l’Ukraine, c’est défendre les Français et les Européens, c’est répondre à une puissance violente qui fait la guerre aux portes de l’Europe, qui multiplie les attaques informationnelles, les cyberattaques et les manœuvres de déstabilisation contre les intérêts

ses actions ont déstabilisé les marchés agricoles comme elles ont déstabilisé le marché de l’énergie. Les céréales ukrainiennes ont perdu leur débouché principal de la mer Noire. Malgré les corridors de solidarité mis en place en Pologne et en Roumanie, avec le soutien de l’Union européenne, un trop grand volume de ces céréales reste stocké en Europe, en particulier dans les États membres frontaliers de l’Ukraine. Dans ce contexte, notre pays – c’est tout à son honneur – a, depuis le début du conflit, soutenu des mesures temporaires facilitant les échanges avec l’Ukraine ; pour autant, solidarité ne signifie pas naïveté.

pour une durée maximale de 120 jours afin de limiter l’impact de la libéralisation du commerce de ces produits. Vous avez raison de mentionner la situation différente des œufs, des volailles et des céréales. Nous avons agi sur les deux premiers produits, nous continuons à négocier sur le troisième. La position de la France est sans ambiguïté : nous défendrons nos agriculteurs.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur le projet de Pass Rail à 49 euros qu’avait annoncé votre prédécesseur, en faisant fi des nombreuses alertes du secteur ferroviaire, mais surtout de celles des régions, qui financent les TER.

et que la SNCF présente d’excellents résultats depuis trois années, ce dont nous pouvons tous nous réjouir. Pour autant, il me semble que, en annonçant dans des délais si brefs l’instauration d’un pass à 49 euros calqué sur le modèle allemand, le gouvernement précédent a réalisé une opération de communication sur le dos des régions et de leurs finances. Je l’avais dit à l’époque : cessons d’avoir de bonnes idées avec l’argent des autres ! Il n’a échappé à personne que les régions financent déjà massivement les transports ferroviaires régionaux.

Pour l’ensemble des régions de France, cela représenterait un manque à gagner de 200 millions d’euros, et jusqu’à 950 millions d’euros pour l’Île de France. Comment cautionner une telle utilisation de l’argent public ? Le véritable problème du train en France n’est pas la demande, mais bien l’offre. Monsieur le ministre, dans le cadre de votre prise de fonctions, envisagez vous de reprendre à votre compte cette promesse ou pourriez vous privilégier des aménagements en faveur d’un abonnement plus resserré, notamment en direction de la jeunesse, dont les moyens financiers et de mobilité sont beaucoup plus restreints que ceux du reste de la population ?

vous avez raison, la mobilité est affaire de pragmatisme. Je partage l’idée d’un distinguo à opérer, selon que l’on est confronté à un problème de demande ou d’offre en matière de transport,

qui disposent de compétences étendues en matière de transport et qui pratiquent également des tarifications différenciées. C’est donc avec une forme de pragmatisme et une volonté de travail en commun avec les régions que je souhaite me saisir de ce dispositif. J’envisage

les jeunes et sur la période estivale, pour les réseaux Intercités et TER. Il s’agirait, en quelque sorte, d’une tarification sociale pour les jeunes, afin de leur permettre de découvrir l’ensemble des régions de notre beau pays,

Les Républicains. Informations relatives à l’adaptation au changement climatique, à la pollution, à la gestion des ressources hydriques et marines, à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire informations relatives aux communautés affectées, aux utilisateurs et consommateurs finaux… Voici quelques exemples des nouvelles informations que les entreprises devront fournir pour répondre aux nouvelles exigences de la directive CSRD () que vous avez transposée par ordonnance en décembre dernier.

Comment pensez vous accompagner les entreprises dans ce fastidieux exercice, madame la ministre ? Qui pourra traduire le vocabulaire technique en langage clair, accessible et compréhensible par les dirigeants d’entreprise ? La délégation sénatoriale aux entreprises propose une pause jusqu’à l’application totale de la directive, c’est à dire jusqu’en 2028. Je rappelle que le contenu de la déclaration de performance extra financière a été modifié vingt et une

pour la réplique. Les agriculteurs manifestaient il y a peu contre l’inflation administrative et normative. Faites en sorte que nos PME françaises ne suivent pas le même mouvement, rallongeant ainsi le long cortège des incompris et des mécontents, La parole est à Mme Monique Lubin, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Madame la ministre, la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception prévoit la tenue obligatoire de trois séances d’éducation à la vie affective et sexuelle au cours d’une année scolaire. Ces séances sont essentielles pour prévenir les pratiques sexuelles à risque auprès des jeunes, pour leur permettre de mieux appréhender la notion de consentement et pour les sensibiliser aux violences sexistes ou sexuelles

Et lorsque des établissements se décident à les mettre en place, ils se trouvent de plus en plus souvent sous le feu d’organisations, soutenues la plupart du temps par la droite conservatrice et l’extrême droite, qui contestent par tous les moyens – mise en cause sur les réseaux sociaux, campagnes de désinformation, etc. – la tenue de ces heures dédiées.

La parole est à Mme Laurence Garnier, pour le groupe Les Républicains.

En cette année sportive, il nous semble opportun de profiter de ce moment pour adresser aux femmes un message ferme et clair concernant les principes de la République au regard de la pratique du sport. En France, en 2024, des jeunes filles s’entendent parfois dire qu’elles n’ont pas leur place dans un club de sport parce qu’elles sont des femmes. En France, en 2024, des femmes sont parfois obligées de couvrir tout leur corps à la demande de certains clubs pour pratiquer leur sport. Face à ces difficultés, la loi est confuse. Une petite fille pourra par exemple pratiquer son sport sans voile le mercredi matin dans l’enceinte de l’école et pratiquer le même sport voilée le mercredi après midi dans son club de sport. Madame la ministre, vous avez précisé à juste titre

à toutes les jeunes filles qui ne veulent pas de cette liberté conditionnelle, madame la ministre ? Que faites vous pour protéger les femmes de ces pressions communautaristes et garantir que le sport reste un espace de partage et d’universalisme ?

jamais pour retirer des subventions, des agréments, ni pour fermer des clubs sportifs qui ne seraient pas au rendez vous de la lutte contre le communautarisme et contre le séparatisme. Je suis personnellement allée chercher une cinquantaine de moyens supplémentaires. J’ai formé les fédérations et je leur ai demandé de désigner des référents pour

Il y a quelques jours, le proviseur du lycée Maurice Ravel de Paris a été menacé de mort sur les réseaux sociaux pour avoir simplement rappelé que la loi de la République interdit le port du voile dans l’enceinte scolaire. Lundi, 150 chefs d’établissement se sont rassemblés à la Sorbonne pour soutenir leur collègue. Cette manifestation inédite témoigne du profond malaise qui s’est emparé de l’éducation nationale. Que nous disent ces proviseurs ? Ils nous disent que leur autorité est bafouée au quotidien et que la violence est endémique à l’école. Que les atteintes à la laïcité se multiplient, et qu’elles perturbent désormais la quasi totalité des disciplines. Que beaucoup de professeurs s’autocensurent, car ils ont peur. Ils nous disent que, par aveuglement, angélisme ou négligence, nous payons déjà le prix de nos lâchetés. Ils nous rappellent les meurtres tragiques de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Certains élus de La France insoumise partagent de fausses informations et remettent même en cause la parole du proviseur. Il est inadmissible de mettre sur le même plan la parole d’un enseignant victime de menaces de mort et celle d’élèves qui ne respectent pas la loi. Ces élus jouent avec le feu. Ils sont les complices d’un obscurantisme qui ne cesse de gagner du terrain. En octobre dernier, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, révélait que notre pays compte plus de 1 000 mineurs radicalisés. radicalisés. Certains de ces mineurs radicalisés sont scolarisés sans que leurs enseignants soient informés de leur potentielle dangerosité. Madame la ministre, il est temps de prouver en paroles comme en actes

et inadmissibles. La laïcité est un principe fondateur de notre République. L’article 1 de notre Constitution le dit clairement : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Nous ne pouvons pas tergiverser sur cette laïcité qui est une condition du vivre ensemble. C’est la règle commune à laquelle nous devons tous être attachés, particulièrement dans les établissements scolaires. Je le dis clairement : les établissements scolaires doivent être préservés

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 7 février 2018, on débattait, dans cet hémicycle, d’un projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants. ce texte était de réformer fondamentalement l’enseignement supérieur en modifiant notamment les conditions pour y accéder. À cette tribune, la ministre de l’enseignement supérieur de l’époque avait déclaré que le gouvernement auquel elle appartenait souhaitait, par cette réforme, accélérer accélérer l’élévation générale du niveau de qualification de notre jeunesse, en augmentant le nombre d’étudiants accueillis dans l’enseignement supérieur et en garantissant à tout bachelier le droit d’y poursuivre ses études. Le dessein du Gouvernement était de refonder la « méritocratie républicaine » en donnant à chaque « lycéen où qu’il réside dans notre pays – en métropole ou en outre mer, en milieu urbain ou dans un territoire rural –, les mêmes chances d’aller jusqu’au bout de ses capacités ». Vaste programme

ministre déclarait alors que le principe de personnalisation constituerait un nouvel instrument permettant de rétablir l’égalité des chances au sein de notre enseignement supérieur. Une plateforme informatique, dénommée Parcoursup, devait faire coïncider les choix libres des lycéens et les offres de l’enseignement supérieur. Elle devait garantir l’équité et la transparence des affectations, tout en

Plus qu’un débat technique sur le fonctionnement de Parcoursup, notre groupe a considéré qu’il serait intéressant d’évaluer collectivement les conséquences globales pour les élèves des réformes conjuguées du lycée et de l’accès à l’enseignement supérieur. Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants, nombreux étaient les sénateurs qui avaient dénoncé l’erreur de méthode consistant à réformer l’accès à l’enseignement supérieur avant de modifier substantiellement les modalités de l’examen en

C’est aussi en France que l’écart entre le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement secondaire et celui des diplômés de l’université est le plus important. La situation économique et sociale des individus est fortement déterminée par leur niveau de diplôme, qui est lui même fortement corrélé à l’origine sociale des parents. Cette emprise du diplôme sur les parcours économiques est d’autant plus cruciale en France que l’accès des salariés à la formation professionnelle est restreint. La sélection réalisée au lycée et à l’entrée de l’enseignement supérieur est souvent

avec ses modalités de sélection orientation, ne pardonne guère le faux pas […]. Il amplifie, à chaque étape, les écarts et les faiblesses. Il fonctionne sur l’orientation sélection, peu sur la réorientation. Il est organisé organisé essentiellement par tamis, pas par passerelles. » Reconnaissons objectivement que Parcoursup n’a pas modifié cette situation. Les données collectées après six ans d’application de la réforme montrent que la ségrégation globale à l’entrée de l’enseignement supérieur est demeurée la même.

La Cour des comptes a établi que 20 % des commissions des filières non sélectives, dites « en tension », utilisent le critère du lycée d’origine des candidats. Elles justifient cette pratique par l’importance du contrôle continu dans l’évaluation des résultats des lycéens après la réforme du baccalauréat. On peut se demander si la sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur ne repose pas davantage sur la notoriété des établissements que sur les compétences intrinsèques des candidats.

Je conclurai cette trop rapide introduction en évoquant la situation des bacheliers professionnels. En 2008, dans cet hémicycle, notre collègue Jacques Grosperrin

dont l’essor est maintenant hors de contrôle. Nous partageons toujours l’objectif de la réforme d’accélérer l’élévation générale du niveau de qualification de notre jeunesse. À l’occasion de ce débat, il convient de nous demander si cette ambition a été satisfaite. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, entre les mois de décembre et de juillet, un élève de terminale compose avec un agenda très chargé. En plus des devoirs de fin de semestre, des épreuves anticipées du baccalauréat et du grand oral, nos lycéens sont confrontés aux échéances de Parcoursup : il y a tout d’abord l’inscription, la création du dossier et la formulation des vœux, puis l’arrivée des réponses, les choix et, enfin, la phase d’admission. Pour les lycéens, ce parcours du combattant est crucial, mais combien d’entre eux sont capables de mesurer ce qui se joue pendant cette période ? En décembre dernier, plus de 700 000 familles se sont pressées sur la plateforme pour choisir parmi les 23 000 formations proposées. Selon les chiffres publiés par Parcoursup, 93,5 % des bacheliers ayant émis des vœux ont été destinataires d’au moins une offre d’admission, soit un taux supérieur à celui de l’année passée. Autre évolution positive, les étudiants cherchant à se réorienter disposent désormais de davantage de propositions. qui est de la phase complémentaire, seuls 148 bacheliers sont restés sans proposition. C’est mieux que l’année précédente, mais toujours beaucoup trop pour les familles concernées, et ce malgré l’accompagnement déterminant des élèves sans solution par des commissions d’accès à l’enseignement supérieur

Les choix des élèves sur Parcoursup sont façonnés par des phénomènes d’autocensure et limités par le manque d’information sur les formations. Cette situation n’est pas acceptable. Face à ce constat, je souhaite rappeler les chiffres du sixième rapport annuel du comité éthique et scientifique de Parcoursup (CESP) sur l’offre de formation privée.

Il ne s’agit pas, pour le groupe RDSE, d’opposer l’enseignement public à l’enseignement privé, mais de se demander si les informations dont disposent les jeunes au sujet des différentes formations proposées sur Parcoursup leur permettent de faire un choix vraiment éclairé. Les labels, bien trop nombreux, ne constituent pas une information suffisamment lisible pour les candidats. La charte de Parcoursup prévoit que, en cas d’illégalité, une formation peut voir son référencement sur la plateforme suspendu. Nous appelons à une véritable effectivité des sanctions. Madame la ministre, l’inquiétude dans les foyers, l’angoisse et le stress que peut susciter l’orientation, doivent conduire le Gouvernement à mettre en œuvre des solutions accessibles à tous et compréhensibles par tous, tout en réprimant les fraudeurs et les marchands de rêves. Par conséquent, l’ensemble du groupe RDSE attend vos réponses sur les questions d’accessibilité, de lisibilité et de régulation de la plateforme. La parole

Avant 2018, le dispositif APB était le système principal pour l’admission dans les universités et les écoles post bac. Dans le but de rendre le processus d’inscription plus transparent,

La plateforme est également apparue comme une petite révolution pour les élèves : elle leur a donné une liberté totale dans la formulation de leurs vœux sans avoir à les hiérarchiser – nous savons combien cela leur est cher. Cette évolution a permis de lutter contre l’autocensure dont on mesure à quel point elle peut être forte lorsque l’entourage familial n’est pas sensibilisé au monde de l’enseignement supérieur.

On l’oublie souvent, mais cette mesure, tout comme la valorisation des parcours en cordées de la réussite, est un vrai levier pour lutter contre les inégalités. Cela ne règle pas tout, bien évidemment, mais c’est un progrès que Parcoursup concrétise chaque année. Force est de constater que, dans l’ensemble, malgré les nombreux articles de presse qui portent chaque année sur les soi disant dysfonctionnements du dispositif, les résultats sont au rendez vous. En témoignent les chiffres pour l’année 2023 917 000 candidats étaient inscrits sur la plateforme, et la procédure a permis à 93,5 % des bacheliers d’obtenir une proposition d’admission dans l’enseignement supérieur.

La difficulté du choix fait partie intégrante de l’apprentissage. La limiter est une évidence, la supprimer serait un non sens. Depuis l’avènement de Parcoursup, le Gouvernement n’a eu de cesse d’améliorer le dispositif, tant en termes d’ergonomie que sur le fond, notamment en intégrant de nouvelles fonctionnalités

Cette réforme continue témoigne, madame la ministre, de votre engagement à améliorer constamment le processus d’orientation et d’admission dans l’enseignement supérieur. Tout d’abord, une attention particulière a été portée à l’accompagnement des lycéens tout au long de leurs démarches sur Parcoursup. Des outils interactifs ont été développés pour aider les élèves à mieux comprendre les différentes filières et leurs débouchés professionnels. Des ressources pédagogiques supplémentaires ont également été mises à disposition pour soutenir les lycéens dans leur choix d’orientation. Ensuite, une amélioration significative a été apportée à la transparence des critères d’évaluation des dossiers. Les élèves et leurs familles ont désormais un accès plus simple et plus détaillé aux éléments pris en compte lors de l’examen des candidatures, ce qui leur permet de mieux anticiper les attentes des établissements d’enseignement supérieur. Enfin, des ajustements ont été effectués pour améliorer la fluidité et l’efficacité du processus d’admission. Des améliorations techniques ont été apportées à la plateforme pour garantir une navigation plus fluide et une meilleure gestion des candidatures.

La mise à jour de décembre dernier a par ailleurs rendu plus aisée la comparaison entre les offres, en permettant notamment aux lycéens de mieux s’informer sur le contenu des formations, leur statut, le taux de pression, ainsi que sur les frais de scolarité, ce qui constitue une avancée significative pour rendre le processus d’inscription plus transparent et plus équitable. Je crois comprendre qu’il ne s’agit pas là de l’unique amélioration. Je souhaiterais connaître, madame la ministre, les nouveautés apportées à Parcoursup pour la session 2024. Ces dernières visent elles à répondre aux préoccupations des lycéens et de leurs familles, et à garantir une meilleure orientation des candidats dans l’enseignement supérieur ?

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, qu’il s’agisse des étudiants actuels ou futurs, notre jeunesse est en proie à une forte anxiété. La période du covid 19 l’a profondément affectée et la santé mentale des jeunes de notre pays est devenue une urgence sanitaire. Notre jeunesse souffre aussi d’une précarité grandissante que les files d’attente devant les banques alimentaires nous rappellent quasi quotidiennement. On ne peut pas dire que les annonces de ces dernières semaines soient de nature à rassurer les jeunes : ni l’annonce de près d’un milliard d’euros de coupes dans le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui affectera nécessairement les conditions de la réussite de leurs études,

On est lâchés dans la fosse », m’ont dit les étudiants que j’ai pu rencontrer. Cette anxiété découle d’un mensonge initial : Parcoursup a été présenté comme une réponse méritocratique à l’injustice du système précédent, et la sélection comme un remède à l’échec dans les études supérieures. En réalité, la fonction première de la plateforme a été de gérer la pénurie dans un système universitaire sous financé alors qu’entre 2008 et 2021 le nombre d’étudiants a augmenté de 25 %, le budget de l’enseignement supérieur a quant à lui chuté de 12 %. Parce que l’objectif réel de Parcoursup n’est pas pleinement assumé, la procédure s’apparente pour les candidats à un parcours semé d’embûches, source d’injustices et de défiance. Le dernier rapport du comité éthique et scientifique de Parcoursup, publié lundi dernier, pointe de nouveau les failles du système, en particulier le manque de transparence de la sélection. Les auteurs du rapport regrettent l’opacité des critères quantitatifs utilisés pour le préclassement des candidats par les commissions d’examen des vœux. de certaines formations expliquent tenir compte des spécialités pour classer les candidats, les informations sur la pondération de ces notes sont absentes des grilles d’analyse présentes sur Les candidats ont besoin d’informations claires pour orienter leur choix. Cette transparence est nécessaire pour que les lycéens aient confiance dans la procédure. Or, pour beaucoup d’entre eux, ce n’est pas le cas. Cette situation contribue à la fuite vers les établissements privés qui captent un nombre toujours plus important d’étudiants, alors que les formations laissent souvent à désirer, quand elles ne relèvent pas de l’arnaque. les responsables de chaque formation rendent publique la formule permettant d’établir leur classement pédagogique. Cette approche faciliterait l’acceptation des décisions d’affectation

c’est l’inégal accompagnement dont bénéficient les lycéens face à la masse d’informations présentes sur la plateforme pour détailler les plus de 20 000 formations qui y

les lycéens mettent à mal leur estime de soi. C’est dans cette brèche que s’est engouffré le marché privé de l’accompagnement à l’orientation, dont le recours est socialement et économiquement inégalitaire. Madame la ministre, comment comptez vous renforcer le service public de l’orientation et mieux accompagner les lycéens les moins bien préparés pour faire face au flot d’informations présent sur la plateforme ?

Voilà, je crois, un court, mais parfait résumé de ses défaillances, encore trop nombreuses et criantes. Certes, de nombreux progrès ont été réalisés, à l’instar de l’élargissement de l’offre de formation, de l’enrichissement de l’information ou de l’ajustement du calendrier.

Nous devons donc nous demander pourquoi, malgré les efforts consentis, prédominent dans le débat public une anxiété croissante et le sentiment d’un manque de clarté, d’équité et de transparence. nous demander pourquoi cet outil, présenté comme « une procédure simple, juste et transparente » par Frédérique Vidal et Jean Michel Blanquer, s’assimile désormais de plus en plus à la matérialisation d’un cauchemar annuel pour les élèves et leurs familles. Complexité technique de la plateforme, absence d’examen des lettres de motivation, opacité totale des critères de sélection… Les maux sont connus de tous et leurs conséquences sont de plus en plus préoccupantes. Voilà en effet six ans que les étudiants cherchent des stratégies

Inscrire les heures d’orientation dans la grille horaire des enseignements et les sanctuariser ; renforcer la formation des professeurs principaux et des référents en matière d’orientation : voilà deux mesures

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à huit jours de la clôture des inscriptions sur la plateforme Parcoursup, débattre de l’équité et de la transparence de cette procédure d’admission dans l’enseignement supérieur prend tout son sens. Force est de constater que, depuis sa création en 2018, Parcoursup n’a jamais suscité la pleine et entière confiance des élèves et de leurs parents : ce dispositif fait l’objet de critiques récurrentes portant notamment sur l’opacité des modalités de classement et sur un certain manque d’équité. Or, sans confiance, il ne peut y avoir d’adhésion. Toutefois, cette défiance repose en partie sur des appréciations infondées. renvoie l’imaginaire collectif, Parcoursup n’examine pas les candidatures des futurs étudiants et ne procède à aucun classement. Ce rôle incombe aux établissements d’enseignement supérieur et aux commissions d’examen des vœux, dont les jurys sont souverains et les délibérations sont confidentielles, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel. L’indépendance des jurys et l’autorité de leurs décisions sont sans conséquence sur la qualité du processus de sélection. Bien entendu, la procédure est perfectible et doit encore gagner en lisibilité et en transparence – les membres des jurys le reconnaissent volontiers. J’ajoute qu’elle doit aussi gagner en rapidité, car la longueur de la procédure et l’incertitude que cela emporte accroissent la défiance vis à vis de ceux qui prennent la décision d’admettre ou non un élève dans la filière de formation qu’il a choisie. Les établissements d’enseignement supérieur sont d’autant plus incités à parfaire leur processus décisionnel que ce manque de transparence a été souligné à plusieurs reprises par le Défenseur des droits et la Cour des comptes, mais également par l’inspection générale de l’éducation nationale et le comité éthique et scientifique de Parcoursup.

Dans ce contexte, il me semble extrêmement important que la fiche Avenir renseignée par les lycées soit la plus précise possible – plusieurs présidents d’université m’ont invitée à plaider en ce sens. Celle ci est particulièrement importante, car elle comporte des appréciations pour chaque vœu formulé par le lycéen pour la phase principale.

Par ailleurs, nous pouvons légitimement nous interroger sur l’impact des algorithmes dans l’étude des demandes d’admission. Nous le savons, les universités recourent de manière systématique à un algorithme de préclassement. Dès lors que le traitement informatique est prédominant, comment Parcoursup procède t il pour mesurer le mérite ? Quelle est la place des personnes chargées de la sélection au sein des établissements supérieurs ? Les algorithmes ne doivent pas remplacer l’humain, et l’opacité doit absolument être

Quant aux enseignants, ils en arrivent à ajuster les dossiers scolaires, afin de maximiser les chances de réussite de leurs élèves… Un autre point mérite d’être relevé : les distorsions d’évaluation, que la plateforme ne semble pas être en mesure de pondérer, créent de véritables iniquités.

Le Sénat s’est saisi de ce sujet en juin dernier, en dressant un état des lieux du fonctionnement de la plateforme numérique. Notre collègue Jacques Grosperrin, dans son rapport d’information, a formulé huit recommandations qui pourraient remédier aux failles de Parcoursup. Madame la ministre, si des améliorations ont été apportées à la procédure Parcoursup depuis sa création, de nombreux dysfonctionnements perdurent. Quelle traduction réservez vous aux recommandations émises par Jacques Grosperrin ? Comment entendez vous,, redonner confiance aux élèves et aux parents ? Merci

et d’équité. J’aborderai la question de l’équité à travers trois sujets. Le premier concerne les élèves boursiers. Pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur des élèves des catégories sociales les moins favorisées, la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants a instauré, dans le cadre de Parcoursup, des quotas de boursiers dans les formations non sélectives en tension.

Je vous remercie,

La compréhension et la transparence des algorithmes sont essentielles pour comprendre et faire confiance à un tel instrument, par lequel des décisions déterminantes pour la vie des jeunes sont prises.

Cette lucidité doit se traduire en actes. Parcoursup est à l’image d’une politique et d’un système toujours plus sélectifs et méritocratiques, qui perpétue les inégalités sociales et contredit

entre 1980 et 2022, alors même que le nombre de lycéens, sur cette période, est passé de 1,4 million à 2,2 millions. De plus, le manque de places dans l’enseignement supérieur est très important. Ce qui se joue derrière le budget et les moyens alloués à cette fameuse frontière entre lycée et enseignement supérieur, c’est l’accès de tous les jeunes étudiants à un enseignement supérieur de qualité,

l’existence de règles et du respect de ces règles ». Dès lors, que répondez vous à la grande majorité des lycéennes et des lycéens qui subissent les vœux de Parcoursup alors que, au même moment, des établissements élitistes comme Stanislas, à Paris, contournent sans vergogne la plateforme pour leurs élèves privilégiés ?

Que comptez vous faire concrètement pour agir contre ces inégalités ? Quelles mesures envisagez vous de prendre pour rendre Parcoursup enfin plus transparent et, surtout, plus égalitaire – peu importe que l’on vienne d’un grand lycée parisien, d’un lycée de campagne ou d’une école française à l’étranger –, et pour que les jeunes puissent faire des choix véritablement éclairés pour leur avenir

Mme la ministre.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, convenons en, Parcoursup est un système en évolution,

attirer votre attention sur le fait que, si un grand nombre de bacheliers généraux trouvent effectivement une formation sur la plateforme,

par le ministère du travail, ce qui prête nécessairement à confusion. Ainsi, de nombreux jeunes paient cher ces formations privées pour se retrouver très peu formés. Je sais qu’un groupe de travail ministériel se penche actuellement sur la question de l’enseignement supérieur privé à but lucratif. Aussi, madame la ministre, quelles dispositions envisagez vous de prendre ou de recommander,

La plupart des enquêtes concernant le ressenti de celles et de ceux qui ont utilisé Parcoursup soulignent par ailleurs une certaine opacité quant aux algorithmes de tri et au classement des candidats, accentuant de fait le stress de nos enfants et des parents.

? Surtout, nous devons distinguer l’outil, à savoir la plateforme, du contexte plus général, à savoir la réforme du lycée et des filières universitaires et techniques. La plateforme Parcoursup est en fait un instrument qui combine orientation et sélection. Elle vise à informer le lycéen des différentes possibilités qui lui sont offertes et, donc, à l’orienter dans ses choix. Elle sert aussi, au regard des candidatures, à sélectionner les jeunes retenus dans chaque filière.

Enfin, pourquoi ne pas utiliser en amont de la phase officielle un simulateur reposant sur l’intelligence artificielle ? Il permettrait, à partir des données statistiques des années précédentes et des souhaits génériques du

Mais l’essentiel réside dans l’impact de la réforme du lycée et la programmation des épreuves de spécialité du bac au mois de juillet. Si cette dernière décision a incontestablement des vertus pédagogiques, elle rend les notes du contrôle continu du premier semestre, voire du premier trimestre, plus importantes que celles des épreuves écrites de spécialité du baccalauréat. Cela pose donc la question essentielle de l’homogénéisation des notes entre les différents lycées et, subséquemment, de nouveau la question de l’équité. Je vous invite également à veiller à ce que la réforme du bac ne pousse pas les lycéens à choisir à terme des spécialités leur assurant une meilleure orientation au détriment de celles qui sont pourtant nécessaires à l’exercice des métiers essentiels pour l’avenir de notre pays.

Il est notamment reproché au dispositif un manque de transparence, d’équité, de clarté et de rapidité. Malgré les améliorations apportées à la plateforme, par exemple une offre de formation élargie et une information enrichie, Parcoursup créerait une égalité de façade, et les élèves seraient choisis uniquement en fonction de leurs résultats scolaires. En réalité, les élèves favorisés ont plus de chances d’avoir de meilleures notes et de bénéficier d’un meilleur accompagnement sur la plateforme. Le processus conduit à une sélection permanente, même dans les études non sélectives comme les

préconisé d’avancer la période de hiérarchisation des vœux en attente à la mi juin, afin de réduire le délai d’attente des propositions pour les candidats qui n’en ont pas et d’accélérer la procédure.

tel accompagnement existe, mais il aurait besoin d’être uniformisé et renforcé au niveau national. L’État doit s’affirmer face à l’essor d’un marché privé qui ne fait qu’accroître les inégalités entre les lycéens, seuls les plus favorisés d’entre eux pouvant y recourir. Lutter contre le manque de transparence il est nécessaire d’inciter les responsables des formations à préciser quantitativement les critères définis et utilisés par les commissions d’examen des vœux. Ce défaut de transparence conduit à des effets pervers.

Enfin, il est nécessaire de faire évoluer Parcoursup, afin de mieux intégrer les candidats en reprise d’études. À ce jour, la plateforme est mal conçue pour cette population d’étudiants, qui ne cesse pourtant de croître.

L’enseignement supérieur est libre dans notre pays. Par conséquent, la diversité des formations proposées par des structures privées offre aux étudiants une réelle complémentarité vis à vis de l’enseignement public.

à des améliorations techniques, mais aussi, et surtout, grâce à un travail de terrain. Les évolutions que je défends visent trois objectifs : la transparence, l’équité et l’accompagnement à l’orientation, essentiels pour donner confiance dans ce système d’accès à l’enseignement supérieur, réduire le stress des lycéens et assurer tant l’efficacité de l’orientation que la réussite des étudiants.

Cette année, nous avons renforcé l’information sur les taux d’insertion professionnelle, et nous avons permis aux lycéens de comparer plus facilement les formations entre elles.

faute de régulation suffisante, l’enseignement privé sous contrat est confronté à un certain nombre de dérives. Oui, il est temps d’y mettre un terme. Comment concevoir que des établissements financés à hauteur de 73 % par de l’argent public n’acceptent

le Sénat s’était prononcé en faveur d’un contrôle accru de l’instruction en famille au nom de la lutte contre le séparatisme et de la défense de nos idéaux républicains. Nous avons eu raison de le faire. Faisons preuve aujourd’hui du même courage pour lutter contre le séparatisme à l’œuvre au sein de certains établissements privés sous contrat

Veil. Plusieurs établissements imposent des temps religieux à leurs élèves, comme le catéchisme ou la messe, alors que la loi prévoit leur caractère optionnel. Si les langues se délient peu à peu, l’omerta reste de mise, frappant aussi bien les équipes éducatives que les élèves ou les parents. « pas de vague à la puissance 10 », pour citer un professeur exerçant dans le privé. Il est nécessaire de mieux objectiver l’ampleur de ce phénomène, en commençant tout étendre le système de signalement d’atteinte à la laïcité. Récemment interrogé à ce sujet, le ministère de l’éducation nationale a réaffirmé que seul le secteur public était concerné par ce dispositif. obliger les chefs d’établissement de l’enseignement privé à signaler aux rectorats tous les problèmes graves survenus dans leur établissement, ce qu’ils ne sont pas tenus de faire, contrairement à leurs homologues du public, ainsi que le fait remarquer le rapport de la Cour des comptes publié en juin 2023.

Ce montant correspond pour l’essentiel aux rémunérations des 142 000 enseignants, qui sont, rappelons le, des agents du public chargés de délivrer l’enseignement « selon les règles et programmes de l’enseignement public », pour reprendre les termes exacts de la loi Debré.

à rémunérer les personnels non enseignants et à financer les dépenses de fonctionnement, et ce alors que les communes ne disposent pas toujours d’une visibilité sur la façon dont ces fonds sont utilisés, en dépit des dispositions prévues par les textes.

Insuffisamment associés, les rectorats se retrouvent contraints d’accepter des ouvertures de classes, qui leur semblent difficilement compréhensibles au regard de l’évolution de l’effectif global des élèves. À l’heure où les mobilisations se multiplient partout en France pour lutter contre les fermetures de classes dans les établissements publics, ce fonctionnement n’est pas acceptable. On nous reproche toujours, lorsque nous mettons en cause l’enseignement privé sous contrat, de vouloir déclencher de nouveau la guerre scolaire.

Je ne reviens pas sur le sort longtemps réservé au rapport de l’inspection générale sur Stanislas, car le problème ne se limite pas à ce seul établissement. Même lorsque les inspections ont lieu, quelle garantie avons nous que les rapports soient lus et, surtout, pris en compte ? Une fois de plus, l’enseignement privé ne semble pas soumis aux mêmes obligations que l’enseignement public.

soit 23 points de plus que dans le public, et de moins en moins d’élèves de milieux défavorisés. Cette ségrégation rejaillit en miroir sur l’enseignement public. Pour citer le seul exemple de Paris,

Là encore, la Cour des comptes appelle à mieux prendre en considération la composition sociologique et le niveau scolaire des élèves accueillis pour définir les moyens alloués par l’État. Madame la ministre,

la liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. Il en résulte que, si l’organisation d’un enseignement public gratuit et laïque est évidemment un devoir de l’État, cela ne saurait exclure l’existence de l’enseignement privé, non plus que l’octroi d’une aide de l’État à celui ci. C’est ce qu’a indiqué le Conseil constitutionnel dans une décision bien connue

liberté d’enseignement existe, mais cette liberté n’est pas absolue : elle s’exerce, bien entendu, dans le respect de la Constitution, de la loi et de principes essentiels, tels que celui du droit de l’enfant à l’instruction. Le contrôle des établissements ayant passé un contrat avec l’État est ainsi prévu par le code de l’éducation et s’exerce sur le plan tant pédagogique que financier. Alors que des financements publics profitent à l’enseignement privé sous contrat et que les enseignants y sont dans leur immense majorité des agents de l’État, il est en effet normal que ce dernier veille à ce que les engagements pris soient respectés. Au cours des dernières années, nous avons souhaité renforcer ce contrôle sur les établissements privés sous contrat, afin d’en assurer l’effectivité. Cela était, me semble t il, attendu,

est assuré par des hommes et des femmes qui veillent d’abord au respect des exigences pédagogiques. Celles ci doivent être évaluées dans des conditions comparables à celles qui existent pour l’enseignement public.

Nous sommes, de manière générale, particulièrement attentifs au bien être et à l’épanouissement des élèves, dans l’enseignement tant public que privé ; en ce sens, l’enseignement privé doit aussi agir en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement. En un mot, nos inspecteurs s’assurent que le contrat soit bien respecté, et je tiens d’ailleurs à saluer ici leur engagement. Ce contrôle par la puissance publique est d’autant plus nécessaire que l’enseignement privé bénéficie lui aussi de financements de la part de l’État.

de l’État représentaient 55 % des ressources financières des écoles privées du premier degré et 68 % de celles des écoles du second degré. En comparaison, 59 % des financements des écoles primaires publiques et 74 % de ceux des collèges et lycées publics proviennent de l’État.

les aides directes aux élèves, comme les bourses et le forfait d’externat, ou encore certaines dépenses de fonctionnement. Le financement des établissements privés fonctionne selon un principe de parité dit «

Nous veillons de près à ce que ces fonds publics soient utilisés uniquement dans l’intérêt des élèves et dans le respect absolu des principes de la République.

est essentiel, car la France reste l’un des pays de l’OCDE où les déterminismes sociaux pèsent le plus sur la réussite scolaire des élèves. Enfin, disons le clairement, contrairement à ce qui peut être lu ici ou sous entendu là, l’État ne favorise pas l’enseignement privé par rapport à l’enseignement public. J’en veux pour preuve l’ensemble des actions et des indicateurs que nous mettons en œuvre : citons par exemple l’amélioration constante de la qualité de l’encadrement dans le secteur public, sous l’effet des politiques volontaristes menées par le Gouvernement et la majorité, ou encore le développement d’offres de formation attractives dans de nombreux établissements publics, notamment dans des secteurs défavorisés, ce qui permet de faire progresser l’IPS des établissements

Une note d’analyse de France Stratégie révélait récemment : « Dès la petite enfance, on observe une empreinte massive des caractéristiques “héritées” sur les acquis et les performances, empreinte que n’effacent ni l’accueil des jeunes enfants ni le passage par l’école primaire. Au collège se produisent les premières bifurcations de trajectoires. Puis les orientations en fin de troisième amplifient [l]es divergences. […] Aux inégalités d’accès et de niveau de diplôme se superposent au lycée des inégalités liées à la nature et aux spécialités des formations, dont les choix sont eux mêmes fortement dépendants de l’origine sociale et du genre Si l’enseignement privé sous contrat doit justifier en toute transparence l’utilisation des subventions ou du forfait d’externat, par la mise en place d’une comptabilité analytique spécifique, par l’obligation de faire valider ses comptes par un commissaire aux comptes ou encore en communiquant l’ensemble du bilan et du compte d’exploitation à la préfecture pour publication, son implication dans la mixité sociale ne paraît pas aujourd’hui soumise à de tels outils de contrôle ou d’évaluation. S’il est vrai que certains établissements privés sous contrat font le choix d’une forme d’élitisme, au même titre d’ailleurs que certains établissements publics, la grande majorité d’entre eux s’implique fortement dans cette volonté d’accueil de tous, voire des plus fragiles. Pour avoir été secrétaire général d’un lycée privé sous contrat pendant trente ans, je sais combien cette volonté est nationale et s’inscrit dans le projet pédagogique de l’immense majorité des établissements. Ma question, madame la ministre, est donc simple : comment agir pour que la mixité sociale soit une réalité et comment proposer des critères objectifs, qui permettront une plus grande transparence des efforts des uns et des autres dans cette démarche d’accueil de tous nos jeunes ? La parole est à Mme la ministre.

plusieurs axes, dont les trois principaux sont : améliorer l’information des parents d’élèves sur les caractéristiques des établissements privés sous contrat ; renforcer la mixité sociale, en en favorisant notamment la modulation des tarifs en fonction des revenus des parents – 50 % des établissements relevant de l’enseignement catholique devront ainsi proposer sur cinq ans des tarifs modulés – ; enfin, renforcer l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous aurons les premiers résultats de ce protocole au mois de septembre prochain, comme le Sgec s’y est engagé. En outre, la méthode d’allocation des moyens publics aux académies en matière d’enseignement privé est fondée sur la prise en compte des taux d’encadrement, des évolutions d’effectifs

alarmant : les mécanismes de contrôle de l’État sont pour le moins limités, voire inexistants. J’évoquerai à ce titre les trois types de contrôle. Tout d’abord, le contrôle financier de l’État, censé être assuré par les directions départementales et régionales des finances publiques, est pointé du doigt, car il est largement inappliqué. Rares sont les établissements qui adressent leurs comptes aux directions territoriales des finances publiques

du public, représentent 17 % des enseignants sous contrat, mais ils sont rarement inspectés, ce qui compromet la qualité de l’enseignement dispensé. Par ailleurs, aucun inspecteur du second degré n’est chargé de vérifier les emplois du temps des élèves. Enfin, le contrôle

dernier point : la Cour des comptes note que le suivi des contrats se révèle peu rigoureux, certains rectorats ne possédant même pas les documents sur la base desquels les sommes, pourtant importantes, sont versées. Madame la ministre, le Gouvernement doit mettre en œuvre, à l’échelon des rectorats, un programme de contrôle des établissements sous contrat, en lien avec les directions régionales ou départementales des finances publiques. De surcroît, les responsables de l’enseignement privé se montrent favorables au contrôle prévu par la loi.

je précise que nous avons élaboré un vade mecum pour donner des éléments très précis à nos corps d’inspection, afin qu’ils puissent effectuer très concrètement ces contrôles. Enfin, le contrôle administratif est également mis en œuvre de manière progressive. Comme je vous le disais tout à l’heure, il faut sans doute faire monter en puissance l’ensemble

ou tout blanc. Madame la ministre, pour ma part, je n’ai jamais conçu les différentes formes d’enseignement comme une menace pour l’enseignement public, tant je suis convaincu, comme Victor Hugo en son temps, de la hauteur du principe républicain de la liberté d’enseignement, à condition

une certaine caricature et de réaffirmer enfin avec force le principe fondateur de la liberté d’enseignement ? Ne serait il pas temps d’étudier avec objectivité les modalités de réussite de l’enseignement privé sous contrat ? Alors, sans idéologie ni dogmatisme, nous y trouverions peut être quelques clés qui pourraient profiter à notre enseignement public.

Il se trouve que, ayant été rectrice de l’académie de Toulouse, j’ai pu aussi mesurer la diversité des situations, tant dans l’enseignement public que dans l’enseignement privé. Il est vrai que certains établissements privés

en tenant compte des spécificités de chaque régime, mais en veillant à ce que les élèves bénéficient des meilleurs enseignements possible.

Claude Lermytte. Madame la ministre, lorsque des enfants sont scolarisés dans une école privée sous contrat d’association, la commune a l’obligation de participer aux dépenses de fonctionnement de l’école. Le principe de parité entre l’enseignement privé et l’enseignement public mentionné à l’article L. 442 5 du code de l’éducation implique la prise en charge obligatoire des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles des établissements d’enseignement privé sous contrat « dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public

Annuellement, le forfait s’élève donc à 100 000 euros, alors que la commune dispose d’un budget de 500 000 euros ; cela se passe de commentaires… Je tiens également à souligner le grand changement opéré en matière de finances publiques depuis la fixation de l’obligation de scolarisation dès l’âge de 3 ans. Jusqu’en 2019, le forfait communal était appliqué pour les seules classes élémentaires. L’intégration des classes maternelles a fait s’envoler le montant du forfait et les communes, en particulier les plus petites, se trouvent dans une situation budgétaire fragilisée et de moins en moins soutenable. Aussi, madame la ministre, envisagez vous de modifier les règles de participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat accueillant des enfants résidant dans leur territoire ? Quelles mesures comptez vous prendre pour garantir véritablement le respect du principe de parité dans le calcul du forfait communal ? Mme la ministre.

La participation de la commune est calculée par élève et par an, en fonction du coût de fonctionnement relatif à l’externat des écoles publiques ; en cas d’absence d’école publique dans la commune, sa contribution est égale au coût moyen dans les classes publiques du département. Il me paraît important de préciser que seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte et non les dépenses d’investissement, qui, vous le savez, sont exclues du forfait communal. Il appartient aux communes de rappeler ces règles et ces principes aux établissements privés sous contrat qui souhaiteraient obtenir des financements plus plus importants que ceux qui sont prévus par les textes. Je rappelle également que c’est la collectivité qui fixe, par une délibération, le montant du forfait, conformément à la loi. Il existe donc une délibération

les communes, à condition que celles ci puissent justifier d’une augmentation des dépenses et du nombre d’élèves. L’instruction des demandes est faite par les rectorats.

à 73 % par l’État. Ils bénéficient également du financement des collectivités territoriales. Un élève dans le privé sous contrat est source d’économies pour les comptes publics. Comment ? Dans le premier degré, l’élève du privé coûte à l’État 55 % du coût d’un élève du public et, dans le second 68 %. Outre ce constat, des inégalités importantes de moyens persistent entre le public et le privé sous contrat. Si certaines peuvent s’entendre, d’autres ne sont absolument pas acceptables, d’autant qu’elles peuvent avoir des conséquences graves sur l’élève et sa santé. Plusieurs chefs d’établissements vendéens m’ont récemment fait part des difficultés qu’ils rencontrent. Je vous livre un exemple : un élève du public ayant besoin de faire un bilan psychométrique sera pris en charge par le psychologue scolaire. Dans le privé sous contrat, sa famille devra débourser entre 300 et 400 euros. Ce coût pousse certaines familles à y renoncer. Plus largement, en 2011, lors de son audition par la Cour (Dgesco) a reconnu qu’en matière de médecine scolaire l’enseignement privé sous contrat constituait une sorte d’« angle mort des politiques publiques

Alors que 2 millions d’élèves sont scolarisés dans l’enseignement privé sous contrat, devrons nous attendre dix ans de plus avant d’obtenir des données consolidées sur la prise en charge de leur santé ? Comment le ministère compte t il enfin répondre à cette distorsion et rééquilibrer les moyens d’accompagnement alloués à la santé scolaire dans les établissements privés sous contrat ? La parole est à Mme la ministre.

Les obligations de l’État concernant la médecine scolaire sont fixées par la loi. La mission de protection et de promotion de la santé en milieu scolaire incombe au ministère de l’éducation nationale. En l’absence de distinction entre les établissements publics et privés, les élèves qui sont inscrits au sein d’un établissement privé sont également inclus dans ce dispositif global de promotion et de protection de la santé en milieu scolaire, au même titre que les élèves des établissements publics. Par ailleurs, la circulaire du 12 janvier 2001 relative aux orientations générales pour la politique de santé en faveur des élèves, qui a pour objet de fixer le cadre de cette politique, prévoit une application à l’ensemble des élèves scolarisés dans les écoles, les établissements publics d’enseignement, (EPLE) et les établissements privés sous contrat. Le recteur doit définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre de cette politique dans son académie, en tenant compte des axes définis à l’échelon national et, bien sûr, du contexte local. Bien évidemment, des personnels médicaux de l’éducation nationale interviennent ponctuellement dans les établissements privés sous contrat, notamment dans le cadre des bilans obligatoires, des campagnes de vaccination obligatoire ou bien à la demande des chefs d’établissement en cas de difficulté particulière nécessitant l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire. Les établissements privés Les établissements privés sous contrat peuvent toutefois disposer de personnels médicaux de droit privé, sur lesquels nous n’avons pas de visibilité. Pour être parfaitement honnête avec vous, madame la sénatrice, j’ai actuellement en

d’abord fallu la résolution personnelle d’un ancien ministre de l’éducation, Pap Ndiaye, pour mettre en place une enquête administrative. Est il d’ailleurs pertinent que cette décision d’enquête dépende du ministre lui même, alors qu’il existe 4 870 écoles privées sous contrat et 2 870 établissements secondaires, qui nécessiteraient des contrôles ? Il aura fallu ensuite la scolarisation des enfants de la ministre de l’éducation dans ce même établissement. Il aura fallu enfin un enchaînement médiatique et la publication du rapport d’inspection, par voie de presse

Aussi ai je demandé à la commission de la culture du Sénat une commission d’enquête visant à mesurer l’efficacité du contrôle de l’État sur le respect des obligations des établissements scolaires privés sous contrat.

professeure de droit public que vous êtes. L’article 1 de la loi Debré éclaire la situation : « L’établissement sous régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, propre, doit donner son enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. » Ces dispositions sont reprises à l’article L. 442 1 du code de l’éducation, selon lequel l’enseignement est dispensé « selon les règles et programmes de l’enseignement public La difficulté d’ordre juridique et presque philosophique réside dans l’articulation entre les obligations de service public et cette notion de « caractère propre », qui n’est pas définie par la loi. L’enseignement catholique, dans son statut de 2013,

Certains établissements confessionnels demandent même aux parents de signer une charte par laquelle ils acceptent que « le message de l’Église catholique soit présenté et promu comme chemin de croissance et de vérité auprès des élèves ». complètement incluse dans le cursus et présentée comme comparable aux enseignements sur le fait religieux du programme national, qui sont fondamentalement critiques, au sens de la critique historique. Ma question, peut être un peu complexe, madame la ministre, est la suivante : comment pouvez vous nous garantir que le « caractère propre » de ces établissements n’entre pas en conflit avec le respect de la laïcité et de la liberté de conscience des élèves et des enseignants ? Pouvez vous nous donner l’assurance que l’État ne subventionne pas des tâches relevant du caractère propre de l’établissement, ce qui entrerait en totale contradiction avec le principe de la séparation des Églises et de l’État ? Monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias, vous le savez, la liberté de l’enseignement est un principe à valeur constitutionnelle, qui fonde l’existence de l’enseignement privé. Le caractère propre des établissements privés, notamment pour ceux qui revendiquent un caractère propre confessionnel, est bien reconnu par la loi. L’article L. 442 1 du code de l’éducation, que vous avez cité, y fait référence, en établissant que les établissements scolaires privés sous contrat, tout en conservant leur caractère propre, sont tenus de faire preuve d’une certaine neutralité et doivent respecter les programmes de l’éducation nationale et les valeurs de la République. Je le dis ici clairement, les valeurs de la République sont premières ; le caractère propre est un élément qui caractérise l’établissement, mais, au sein de celui ci, les valeurs de la République sont premières. Très bien ! Les écoles et les établissements scolaires privés sous contrat sont donc tenus de faire partager à leurs élèves les valeurs de la République, parmi lesquelles figure la laïcité, que les élèves de tous ces établissements doivent apprendre à respecter. Peuvent s’y ajouter des options autour de ce que le caractère propre d’établissement confessionnel peut porter. La loi du 2 mars 2022, qui vise à combattre le harcèlement scolaire, a désormais inscrit à l’article L. 111 6 du code de l’éducation une obligation de moyens de lutte contre le harcèlement dans tous les établissements d’enseignement privé cela a à voir avec ce dont nous parlons. De manière très concrète, le double respect du caractère propre de l’établissement et des valeurs de la République conduit par exemple à ne pas imposer l’affichage de la charte de la laïcité dans les les établissements privés sous contrat, puisque cela relève de la vie scolaire. Toutefois, les établissements doivent respecter, je le répète, les valeurs de la République ; c’est pour moi tout à fait essentiel. En matière de signes d’appartenance religieuse, c’est le chef d’établissement et le règlement intérieur de l’établissement qui pourront être utilisés pour tolérer ou, au contraire, prohiber certains signes en fonction du caractère de l’établissement. La parole est à M. Bernard Fialaire.

la question de ce qui relève du caractère propre d’un l’établissement. Le ministère a diffusé à l’ensemble des réseaux d’enseignement privé sous contrat des recommandations pour organiser un temps de recueillement et d’hommage à Dominique Bernard, comme dans les établissements publics. Toutefois, en vertu de leur caractère propre, les établissements privés sous contrat peuvent bien entendu s’exprimer librement sur tout ce qui ne relève pas du strict respect des programmes scolaires ou des valeurs de la République.

peut être la ligne de partage. Les écoles et établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, sont évidemment tenus de faire partager à l’ensemble de leurs élèves, je l’ai dit tout à l’heure, les valeurs de la République,

par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement de l’externat des écoles publiques. Je l’ai dit précédemment et je le répète, seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte, non les dépenses d’investissement. Par ailleurs, les avantages consentis par les collectivités pour le fonctionnement des classes sous contrat ne peuvent pas être supérieurs à ceux qui sont consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes de l’enseignement public. Pour répondre directement à votre question, mais également à celle de M. le sénateur Fialaire, s’il est vrai que certaines dépenses sont directement corrélées au nombre d’élèves et de classes,

Mme Catherine Belrhiti. Madame la ministre, le thème du débat de ce jour me touche particulièrement. Ayant enseigné au sein d’établissements privés sous contrat pendant trente cinq ans, j’en connais les avantages et les inconvénients, tout comme les critiques dont le modèle peut faire l’objet. Il faut, je le crois, rappeler d’emblée une évidence : l’enseignement privé sous contrat est un acteur essentiel du service public de l’éducation de ce pays. Représentant près de 20 % des effectifs scolarisés, il offre une liberté de choix aux parents qui souhaitent, pour des raisons qui leur sont propres, scolariser leurs enfants dans un établissement plutôt que dans un autre. Notons que la proportion d’enfants scolarisés dans le privé est stable depuis quelques années, tout comme d’ailleurs le financement de ces établissements. Le débat, à mon sens, porte donc non pas sur les moyens investis par l’État, mais véritablement sur les obligations qui incombent à ces établissements, en contrepartie de ces moyens. J’insiste souvent, au sein de la commission de la culture et de l’éducation, sur le fait que, en tant que citoyens français, nos droits sont nécessairement complétés par des devoirs. C’est là, je le pense, la condition du maintien de notre équilibre démocratique et social. La situation de l’enseignement privé sous contrat doit s’analyser au travers du même prisme. La loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, n’a cherché ni à priver l’État d’un droit de regard ni à priver les établissements privés de devoirs. L’objectif du contrat d’engagement était au contraire de dégager un compromis permettant de maintenir la liberté d’enseignement tout en instaurant un véritable contrôle de l’État. À l’aune de ce débat, c’est bel et bien ce contrôle qui semble défaillant. À la suite des récents événements, je vous demande donc, madame la ministre, quelles mesures entend prendre concrètement pour renforcer le contrôle des établissements privés sous contrat, afin de les maintenir dans le cadre légal et les valeurs instaurées par la loi Debré.

La proportion d’élèves très favorisés dans les collèges privés est de 40 %, soit le double de ce qu’elle est dans le public. L’écart s’est creusé de près de dix points en vingt alors même que les effectifs sont stables. La part des élèves boursiers dans le secondaire est trois fois plus faible dans le privé que dans le public. Il y a là un véritable séparatisme, contre lequel nous devons lutter avec acharnement. Pis, une étude de 2014 menée par trois chercheurs au moyen d’une expérience contrôlée, inspirée de la méthode du, a démontré qu’il existe à l’entrée des établissements scolaires privés une sélection ethnique. Malgré tous les protocoles, rien ne change. De fait, nous n’avons pas, aujourd’hui, les moyens de savoir comment les établissements privés sélectionnent leurs élèves ni de contrôler les efforts qu’ils font, ou pas, en faveur d’une plus grande mixité. l’application Affelnet ou la mise en place d’une plateforme d’inscription dans les établissements privés, à l’entrée en sixième et en seconde, permettrait d’avoir des données précises sur le profil des élèves qui se portent candidats et sur celui de ceux qui sont effectivement retenus par les établissements privés. telle plateforme donnerait aussi les moyens à l’État de contraindre l’enseignement privé sous contrat à respecter ce contrat, en accueillant tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance. Madame la ministre, Madame la ministre,

d’ailleurs savoir que certains établissements ont été condamnés pour avoir refusé d’accueillir des élèves qui présentaient un profil

Mme Anne Ventalon. Madame la ministre, au mois de décembre dernier, Gabriel Attal annonçait, pour la rentrée 2024, la mise en place de trois groupes de niveau en français et en mathématiques pour les élèves de

près de 20 % des élèves. Seule la suppression de l’heure de sixième actuellement dédiée à l’approfondissement du français et des mathématiques contribuera au financement, ce qui est loin de couvrir les besoins. ce sont donc les moyens ordinaires consacrés par le privé à la création d’options ou de filières ou à des ouvertures de classes qui devront être utilisés ; voilà qui n’est pas acceptable. Madame la ministre, comment financerez vous les groupes de niveau dans le privé ? vigueur de la loi dite Debré de 1959, les chefs d’établissement et leurs équipes définissent ensemble leur organisation et un projet éducatif spécifique, pourvu qu’ils respectent les programmes de l’éducation nationale. concerne les groupes de niveau, les établissements semblent donc les mieux à même de définir leurs besoins. Je rappelle que, dans le privé sous contrat, les collégiens en difficulté en français représentent 15 % des effectifs de contre, dans le public, 25 % hors éducation prioritaire et 52 % en éducation prioritaire renforcée. On ne saurait donc appliquer la même règle à tous. Aussi ma deuxième question est elle la suivante : les établissements privés sous contrat conserveront ils, en vertu du principe d’autonomie, leur liberté de choix dans l’application de la réforme ? La parole

privé ou public, une ambition, celle d’élever le niveau scolaire de nos élèves. Nous considérons qu’à cet égard la possibilité de travailler en groupe, en sixième et en cinquième, sur les matières fondamentales que sont le français et les mathématiques

des collectivités territoriales, à des degrés divers, selon la forme du contrat, aux dépenses de fonctionnement. Mais il impose aussi des devoirs, en particulier celui de dispenser les enseignements par référence aux règles et aux programmes de l’enseignement public, ou encore celui d’accueillir les enfants sans distinction d’origine, d’opinion

à ces engagements puissent être identifiés et signalés, dans le privé comme ailleurs. Madame la ministre, vous avez plusieurs fois fait état, durant ce débat, des moyens dont dispose votre ministère pour effectuer ces contrôles selon une périodicité raisonnable.

est plutôt de savoir si l’engouement croissant pour les écoles privées, dont nous parlons depuis l’ouverture de notre débat, n’est pas le miroir des faiblesses actuelles de l’école publique. ! Madame la ministre, tant que l’État n’investira pas davantage dans son école publique, tant que l’on continuera à fermer des classes sans apporter de réponses claires et fermes aux crises successives que vivent trop d’établissements,

quant à elle, ne peut pas se payer le luxe de la guerre scolaire, comme le rappelle souvent Max Brisson ; or toutes les politiques publiques qui s’y rapportent se fondent sur des logiques comptables qui ne tiennent pas compte de ses spécificités.

des établissements neufs, rationalisés, dans lesquels on continue pourtant encore et toujours à fermer des classes. Comment, dans ce contexte, ne pas se poser la question de la fiabilité de ce modèle ? En éloignant l’école des habitants, on a petit à petit porté atteinte à la qualité de vie dans nos campagnes et réduit l’attractivité de nos territoires. Afin de répondre aux attentes des Français, qui sont plus attachés que jamais

plus long terme, afin de prévenir les difficultés que vous évoquez. Cela a été dit, au cours des derniers mois, plusieurs dysfonctionnements au sein de certains établissements privés sous contrat ont été mis au jour. Cette réalité ne doit pas être éludée : s’il existe des torts, il faut les redresser, sans tomber dans la caricature ni relancer la guerre scolaire.

Il semble que non ; or, pour beaucoup, cette situation suffit à instruire sans nuance le procès de l’enseignement privé. Pourtant, ses établissements n’ont jamais refusé de se prêter à un tel contrôle, comme l’a récemment rappelé le secrétaire général de l’enseignement catholique.

Or, dans son rapport de juin 2023, la Cour des comptes relevait que ce contrôle reste « largement inappliqué ». Les responsabilités sont probablement partagées, et les établissements qui ne respectent pas leurs obligations doivent être rappelés à l’ordre. Il y a aussi matière, sans doute, à améliorer le recrutement des chefs d’établissement pour le rapprocher des exigences qui prévalent dans le public. Quoi qu’il en soit, il faut traiter les défaillances. Renforcer le contrôle permettra certainement de démontrer aussi que de nombreux établissements peinent à joindre les deux bouts, qu’ils consentent des efforts importants en faveur de l’inclusion et contre le décrochage scolaire, que certains d’entre eux ont déjà créé des caisses de solidarité pour accueillir tous les élèves ou instauré une modulation de la contribution des familles en fonction du revenu des parents pour respecter leurs obligations d’accueil. Au total, le coût pour l’État d’un élève du privé représente la moitié de celui d’un élève du public. Autrement dit, sans les établissements privés sous contrat, la charge publique supplémentaire serait supérieure à 9 milliards d’euros. Le contrôle est la contrepartie de la liberté d’enseignement et de l’autonomie reconnue à ces établissements, qui concourent sans but lucratif au service public de l’éducation.

comme dans de nombreuses communes rurales et de montagne, à Girmont Val d’Ajol, l’école a fermé il y a bientôt vingt ans, et ce malgré l’action des municipalités successives.

: des temps de trajet trop longs peuvent être préjudiciables à la réussite scolaire. Ainsi, madame la ministre, en application du principe de continuité du service public et compte tenu de la nécessité de maintenir une offre scolaire de proximité, ne faudrait il pas envisager d’adapter la carte scolaire aux réalités territoriales, notamment dans les zones de montagne ?

de la CFDT (FEP CFDT) alertait sur la réduction du temps consacré aux disciplines obligatoires au profit d’activités diverses ou à caractère religieux.

la ségrégation croissante dans l’enseignement privé est devenue une sorte de bombe à fragmentation sociale. Absolument ! Alors que la loi Debré précise que tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance, peuvent avoir accès à l’enseignement privé, la ségrégation se renforce. J’y reviens, les chiffres

même que l’enseignement privé sera une fois de plus largement préservé. Pour quelle raison l’enseignement public absorberait il seul la baisse démographique ? Très bonne question ! Je ne vous ferai pas l’injure, madame la ministre, de vous renvoyer à la lecture